L'auteur du débat, en l'occurrence la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, disposera d'un temps de parole de dix minutes, y compris la réplique, puis le Gouvernement répondra pour une durée qui ne devra pas excéder dix minutes.

Monsieur le président, madame la ministre des armées, mes chers collègues, c'est avec gravité que nous abordons le débat de cet après-midi, dans un monde de plus en plus dangereux, où le terrorisme frappe à nos portes et où la guerre est à nouveau possible, du Moyen-Orient à l'Asie nucléarisée, mais aussi aux frontières de l'Europe, avec l'annexion de la Crimée.

pour aller, sans perdre de temps, vers une nouvelle loi de programmation militaire. Au fond, la menace était connue : du terrorisme djihadiste asymétrique jusqu'aux stratégies de puissance dans le haut du spectre- les grandes puissances -, dans un environnement de plus en plus incertain et instable, nous assistions à une accélération de tendances déjà en germe dans le Livre blanc de 2013. La revue remarquablement menée par le député européen Arnaud Danjean confirme pleinement notre analyse. Je voudrais lui rendre hommage personnellement, car il a accepté de consacrer ses compétences, son temps, voire ses vacances d'été, au service de ce devoir important. Il a su réunir autour de lui une équipe compétente et il nous livre aujourd'hui un diagnostic imparable. Mettons de côté les deux composantes de la dissuasion, que le Président de la République lui-même, dans sa lettre de mission, indiquait vouloir maintenir et qui sont donc hors du champ du débat. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées souscrit à cette approche, comme nous l'avons dit dans notre rapport d'information de juin dernier sur la modernisation des forces nucléaires. Ce qui est frappant, c'est évidemment le décalage, le hiatus, pour ne pas dire la contradiction manifeste entre l'aggravation de la menace décrite par la revue stratégique et l'état de nos armées, aujourd'hui saturées d'engagements- je rappelle que plus de 30 000 hommes sont actuellement en opérations intérieures et extérieures -et fragilisées par une décennie d'éreintement et de sous-investissement. Nous en sommes tous responsables

Les crises sont dispersées, depuis les immensités sahéliennes jusqu'à la mer de Chine méridionale et même à l'espace extra-atmosphérique. L'incertitude, la confusion, les menaces hybrides, les postures d'ambiguïté stratégique sèment le doute partout, répandant ce « brouillard de la guerre », parfois jusqu'au coeur de nos alliances. La menace se numérise : cyberattaques sur nos économies et sur nos systèmes politiques, guerre informationnelle et bataille de la communication. Nos engagements, enfin, sont écartelés entre un temps politique précipité par la pression médiatique et un temps des opérations, lequel se compte en années, voire en dizaine d'années. Si la revue n'adopte pas d'approche géographique, une priorité euro-méditerranéo-sahélienne se dessine toutefois, avec une attention particulière portée à notre voisinage immédiat, en particulier à la rive sud de la Méditerranée. Nous y souscrivons pleinement : le danger n'est pas loin. Que se passerait-il si un pays à nos rives était déstabilisé ? Cette revue stratégique doit nous inciter à y réfléchir plus activement. Forts de ce constat, c'est maintenant vers l'étape d'après que nous devons nous tourner : la préparation de la loi de programmation militaire. Or l'état des armées offre, en comparaison, un singulier contraste. Le maintien d'un modèle d'armée complet et équilibré, prôné par la revue, implique, il faut le mesurer pleinement, un considérable effort sur les moyens, car le modèle est bon, mais il est exsangue Trente capacités sont nécessaires pour assumer les cinq fonctions stratégiques. Le maintien de certaines d'entre elles est un défi, la revue le dit sans détour : entrer sur le champ de bataille en premier et durer, en particulier. Entrer en premier sur un théâtre d'opérations, c'est pouvoir agir seul, contre tout type d'ennemi, c'est avoir la capacité d'agréger des alliés, c'est conserver son autonomie stratégique. seulement de combler nos lacunes capacitaires bien connues- moyens de surveillance, ravitailleurs, hélicoptères, moyens de transport stratégique ... -, mais aussi de mener une action réparatrice de régénération du potentiel et d'intégration de l'innovation pour conserver notre ascendant sur l'ennemi.

la force opérationnelle de l'armée de terre entrerait tout entière dans le Stade de France, elle compte moins d'effectifs que la RATP ! Les véhicules de l'avant blindé ont quarante il faudra attendre 2028 pour doter tous les fantassins de leur nouveau fusil d'assaut ; quant au pistolet automatique de l'armée de terre, il a soixante les pilotes d'hélicoptères de l'ALAT, 20 % d'entre eux ne sont pas aptes aux « missions de guerre », faute d'heures de vol. Le format de la marine nationale a fondu ; le programme de frégates multi-missions n'atteindra même pas la moitié de sa cible initiale. Pendant ce temps, la Chine produit chaque année l'équivalent du quart de la marine française. Les pétroliers ravitailleurs, d'âge canonique, ne sont pas aux normes environnementales, les patrouilleurs outre-mer, désarmés, ne sont pas remplacés les hélicoptères Alouette volaient déjà à l'époque de ! Les vingt avions de combat de l'armée de l'air engagés en opérations consomment à eux seuls le potentiel de cinquante appareils

c'est leur compétence qui font la différence dans l'affrontement des volontés que constitue la guerre. Je salue également l'effort et les sacrifices consentis par leurs familles. Dans ce contexte, la remontée en puissance des moyens est indispensable. C'est tout l'enjeu de la prochaine loi de programmation militaire. Le Sénat avait chiffré en juin dernier à 2 milliards d'euros et 4 500 recrutements

d'une décennie de déconstruction. Mais quel paradoxe ! On nous fait miroiter une magnifique remontée en puissance, il ne s'agira en fait que d'une « simple » consolidation. Pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'il faut payer les ardoises du passé.

Et ce n'est pas fini ! Quand les 700 millions d'euros restant seront-ils dégelés ? Qui va payer les 360 millions d'euros d'opérations restant à couvrir pour clore le budget de 2017 ? Ensuite, parce que, sous couvert de vertu budgétaire, la loi de programmation des finances publiques organise un véritable transfert de charge vers la défense pour « neutraliser », voire « siphonner » la hausse des crédits annoncée courageusement par le Président de la République. Attention danger ! La « sincérisation des OPEX »- belle expression ... -ou la résorption forcée de la « bosse budgétaire » sont en fait des outils pour vider de sa substance l'effort de défense annoncé par le Président Or la défense, c'est aussi 200 000 emplois, de haute technologie et non délocalisables ; c'est le premier budget d'investissement de l'État ; ce sont des investissements de rupture et d'innovation, qui tirent toute l'économie ; c'est également 14 milliards d'euros d'exportations par an.

Les armées intègrent, forment et remettent sur le marché du travail des jeunes qui trouvent un emploi. Madame la ministre, vous le voyez, il nous reste du travail. Après cette revue stratégique, les choses sérieuses commencent. Vous pouvez Vous pouvez compter sur le Sénat, sur notre vigilance et notre combativité pour ne pas laisser les armées aux seules mains des comptables. Il faut reconstituer une force armée solide et apte à répondre fermement aux désordres du monde. La revue stratégique en démontre la nécessité, mais notre plus forte exigence reste la sécurité de la France

Cette étude avait un objectif : produire une analyse fine et complète de la situation stratégique internationale et en tirer les conséquences pour notre défense. J'ai confié ce travail à un comité d'experts venus de toutes les disciplines et présidé par M. Danjean, qui a abouti à cette revue stratégique à la fois lucide et ambitieuse pour nos armées, fixant un cap clair et une vision pour la prochaine loi de programmation militaire. Dans quelques instants, je répondrai aux questions que ce document pose sur notre environnement stratégique et l'avenir de notre défense. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir le faire par ces échanges que vous avez voulus plus libres et plus francs et qui permettront d'aborder vos interrogations- celles de la représentation nationale -sans tabou ni fausse pudeur, ce qui est précisément l'objectif de la revue stratégique. Ce travail était un exercice ambitieux.

La revue stratégique fait d'abord un constat : aujourd'hui, la France est plus sollicitée et plus engagée qu'elle ne l'a été depuis longtemps. La menace du terrorisme djihadiste reste centrale pour notre sécurité. Nos ennemis ont changé d'organisation, de visages, de noms, mais ils sont encore plus violents et peut-être encore plus déterminés. Ne nous y trompons pas, la prise de Raqqa et la défaite, sans doute très proche, de Daech ne signifient pas la fin du terrorisme, de son idéologie et de sa barbarie. À cette menace s'ajoute une instabilité croissante aux portes de l'Europe. J'ai à l'esprit les vulnérabilités persistantes dans le Sahel, la déstabilisation durable du Proche et du Moyen-Orient ou la crise migratoire, mais aussi des phénomènes plus larges qui nous touchent et qui appellent le monde entier à s'adapter : les risques pandémiques, les dérèglements climatiques, les trafics ou la criminalité organisée.

Nos armées sont très sollicitées, à l'extérieur comme sur le territoire national, avec pour conséquence une forte mise sous tension de nos capacités et de nos ressources. La revue stratégique, ensuite, prend acte de ce que nous soupçonnions déjà : l'équilibre du monde tel que nous le connaissions à la sortie de la guerre froide est révolu. L'environnement stratégique est aujourd'hui articulé autour de multiples pôles dont les équilibres, les forces et les intentions sont changeants et parfois imprévisibles. Chaque État cherche à affirmer sa puissance, notamment militaire, et entre dans une logique de compétition pour l'accès aux ressources, pour le contrôle des espaces stratégiques et pour l'armement. C'est l'objet d'un troisième constat dressé par la revue : nos forces sont plus contestées et nos ennemis plus équipés et mieux armés.

sont devenus des domaines d'affrontement à part entière, impliquant des acteurs parfois inconnus ou intraçables, dont les actes peuvent avoir des conséquences dramatiques sur notre sécurité et sur le quotidien de nos concitoyens. Enfin- c'est le quatrième constat issu de la revue stratégique -, les nouvelles technologies ont radicalement changé nos forces et nos vulnérabilités.

Cependant, la révolution technologique est aussi un enjeu, car nous devons la saisir pleinement, sous peine d'être dépassés. Enfin, elle peut également devenir une source de vulnérabilité. C'est pourquoi l'espace numérique, dans son ensemble, doit se trouver au centre de nos priorités. Dans cet environnement stratégique à la fois instable et imprévisible, la France est et restera une puissance majeure. Elle continuera à intervenir partout où ses intérêts sont menacés. Sa voix sera entendue, écoutée et respectée. Notre autonomie stratégique n'est pas négociable. Nous la consoliderons, notamment en renouvelant les deux composantes de la dissuasion nucléaire. Nous poursuivrons nos efforts en faveur du renseignement et nous renforcerons de front les cinq fonctions stratégiques : dissuasion, prévention, protection, intervention et connaissance et anticipation, en prêtant une attention particulière à la prévention des risques et des conflits. L'assurance de notre autonomie stratégique passe également par un modèle d'armée complet et équilibré. C'est le gage de notre souveraineté comme de notre liberté. Nous devons être en mesure de détenir toutes les aptitudes et toutes les capacités pour répondre à toutes les menaces. Nous protégerons et nous garantirons notre autonomie totale dans les domaines de la dissuasion, de la protection du territoire et de ses approches, du renseignement, du commandement des opérations, des opérations spéciales ou de l'espace numérique. Dans les autres champs, nous mènerons les partenariats et les coopérations nécessaires pour assurer la pleine capacité d'action de nos forces. Nous assumerons pleinement notre dimension européenne. Nous avons tout intérêt à ce qu'une défense européenne puisse se construire autour d'intérêts partagés. La France, comme l'a indiqué le Président de la République à la Sorbonne le 26 septembre dernier, sera à l'initiative de cette dynamique. Nous avancerons avec ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent. Nous assumerons également pleinement nos responsabilités au sein de l'OTAN et nous renforcerons nos partenariats bilatéraux partout dans le monde. Quand je parle d'Europe, je pense aussi à notre industrie. Nous devons accompagner et encourager le développement d'une industrie européenne de défense solide et réputée. Plus largement, l'industrie et la recherche doivent être au fondement de notre stratégie. C'est un socle économique puissant, une garantie du succès de nos exportations comme de notre innovation. L'innovation, justement, nous devons la prendre à bras-le-corps, en faire notre force et notre moteur. Je parle d'innovation technologique, de recherche, mais également de cet esprit d'innovation qui doit guider toutes les femmes et tous les hommes de la défense. L'audace doit les accompagner dans leurs décisions, dans la recherche de processus plus efficaces, dans la modernisation de notre action. Cet esprit d'innovation est une condition pour l'attractivité de la défense, pour l'efficacité de nos missions et donc pour la sécurité et la liberté des Français. Cette revue stratégique nous offre un apport immense : identifier nos aptitudes prioritaires et agir, agir vite et fermement.

Par ailleurs, le service national universel est une belle idée, mais les armées ne peuvent pas la porter seules : il n'y a pas de nécessité au titre des seules armées, c'est peut-être une nécessité sociale. Aussi, nous contribuerons, si vous nous y associez, comme vous en avez pris l'engagement, à travailler sur ce sujet. Soyons vigilants à reconstituer une belle armée, dont notre sécurité a absolument besoin

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ainsi que le Président de la République l'avait annoncé le 13 juillet dernier à l'hôtel de Brienne, la revue stratégique examine notre environnement et les menaces auxquelles nous sommes confrontés. Elle s'inscrit d'ailleurs très naturellement dans le sillage du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013. On y retrouve la même volonté de jeter un regard lucide et sans concession, pour reprendre vos mots, madame la ministre, sur un contexte « en dégradation rapide et durable », tout en affirmant notre ambition de maintenir notre autonomie stratégique. Elle dresse le constat d'un durcissement des environnements opérationnels, avec le retour des États-puissance- la Russie -ou la fragilisation croissante de certains acteurs étatiques, ou de l'omniprésence des menaces terroristes ou cyber toujours plus diffuses. S'y ajoutent « des fragilités multiples » : démographie, climat, risques sanitaires, criminalité organisée. On ne peut donc que saluer la volonté de relever le défi pour le quinquennat en cours de conserver un modèle de défense complet et équilibré pour agir et répondre à l'ensemble des menaces. Néanmoins, l'intention affichée par la revue stratégique se heurte à la dure réalité des premières annonces. En effet, comme l'a rappelé le président Cambon, outre la coupe budgétaire de juillet dernier qui a affecté les armées à hauteur de 850 millions d'euros, l'intégration au budget de la défense des mesures de « resoclage » budgétaires des OPEX, qui dépassent les 200 millions d'euros le financement des mesures non prises en compte dans la loi de programmation militaire actuelle, décidées en 2016, à savoir 996 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les coûts à venir engendrés par le renouvellement des deux composantes de la dissuasion nucléaire, ne doivent pas compromettre la poursuite d'autres programmes pour nos armées sur le terrain. Certes, l'orientation de notre budget de la défense est à la hausse, avec une augmentation de 1,8 milliard d'euros pour 2018 et 1,7 milliard d'euros en 2019 et 2020. Mais cette hausse utile se révèle en réalité bien limitée. Je vous remercie, madame la ministre, de nous apporter des garanties sur la question centrale des moyens, point d'inquiétude majeure pour nos armées, mais également, et plus généralement, pour nos concitoyens, car il y va aussi des questions de sécurité intérieure. La parole est à Mme la ministre.

vous avez raison d'appeler mon attention, la vigilance s'impose quant aux décisions qui peuvent se prendre ici ou là. Permettez-moi de profiter des dix-huit secondes qui me restent pour vous dire que les 850 millions d'euros d'annulations de crédits étaient en quelque sorte le prix collectif à payer pour régler un certain nombre d'impasses budgétaires, notamment celle qui portait, par exemple, sur le financement des OPEX, mais pas seulement.

La défense et la sécurité nationale, c'est avant tout des femmes et des hommes qui s'engagent pour notre pays. Leurs engagements impliquent leurs familles, qui en subissent les conséquences de plein fouet. Le récent rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire met en évidence de forts enjeux de fidélisation. Difficulté à concilier vie militaire et vie personnelle, mobilité professionnelle du conjoint, reconversion, lassitude face aux difficultés rencontrées en matière d'hébergement sont autant d'écueils. Je voudrais insister ici en particulier sur la politique immobilière du ministère. Même si les crédits vont augmenter en 2018, le parc est très dégradé, sa maintenance ayant été longtemps sacrifiée pour préserver les dépenses d'infrastructures des grands équipements, des grands programmes d'armement. Le rattrapage doit s'inscrire dans la durée et se poursuivre résolument. Il manque 400 logements de militaires en région parisienne. Les logements sociaux de l'îlot Saint-Germain ne seront que partiellement affectés aux familles des militaires 50 sur 250. C'est insuffisant, d'autant que cet immeuble subit une forte décote, de près des deux tiers de son prix, ce qui représente un préjudice important pour le budget des armées. Dans ce contexte, peut-on se passer

monsieur le sénateur, de pointer du doigt l'une des difficultés sans doute majeures qu'éprouvent les militaires et leurs familles

2018. Par ailleurs, dans le cadre du plan Famille que j'annoncerai prochainement, un chapitre entier sera consacré à la question du logement, tant celle-ci est majeure. Il est vrai que nos emprises ont fait l'objet d'une réorganisation en profondeur en Île-de-France du fait de la mise en service, si je puis dire, du grand ensemble de Balard il y a quelques mois. C'est dans ce contexte que le Val-de-Grâce ainsi que l'îlot Saint-Germain ont été mis en vente, dans des cadres différents. Pour ce qui concerne

Paris. Concernant l'îlot Saint-Germain, c'est-à-dire la seconde fraction, celle-ci sera cédée par morceaux ou par sous-ensembles. Vous avez appelé mon attention sur le fait que des décotes importantes ont été réalisées pour les emprises qui avaient déjà été cédées. C'est en effet un sujet de préoccupation, mais, vous le savez, ces décotes sont aussi la contrepartie d'autres engagements, qui permettent également de récupérer, dans le cadre des emprises cédées, un certain nombre de logements pour nos militaires. Il nous revient de trouver le point d'équilibre entre un prix de cession convenable et un nombre de logements obtenus en contrepartie satisfaisant.

Je tiens, madame la ministre, à saluer la qualité du travail réalisé dans des délais contraints, tout en rattachant cette analyse pointue de la capacité militaire de la France au récent plaidoyer du Président de la République pour une Initiative pour l'Europe, Europe qui est, permettez-moi de le citer, « notre histoire, notre identité, notre horizon, ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir ». Je m'attarderai sur un point précis que je considère comme essentiel, l'Europe de la défense et, plus précisément, le fonds européen de la défense. Oui, les défis à relever aujourd'hui et demain en termes de sécurité et de défense sont multiples et complexes ! Les États membres ne sont pas en mesure de les relever seuls. Et il n'appartient pas à la France de les relever seule Avec l'annonce de la création de ce fonds européen le 7 juin dernier, ce constat est désormais contrarié. Il s'agira dorénavant de coordonner intérêts nationaux et autonomie stratégique, industrielle et technologique de l'Europe, d'offrir à l'ensemble des États membres des ressources militaires communes, ce qui permettra ainsi à l'Union européenne de mettre en oeuvre une véritable politique de coopération en matière de défense. La Commission a annoncé que son financement aurait lieu selon les cycles budgétaires de l'Union européenne et à partir de financements nationaux. Madame la ministre, ma question est simple : pouvez-vous nous apporter des précisions sur le calendrier de mise en activité de ce fonds ainsi que sur les estimations en termes de coûts et d'économies pour notre budget national ? La parole est à Mme la ministre. Vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, l'un des objectifs fixés par le Président Macron lors de son intervention à la Sorbonne est de faire en sorte que l'Union européenne dispose à l'avenir d'un véritable budget commun de défense.

certainement lié à une prise de conscience de l'importance des menaces qui pèsent tout autour de l'Europe pour avancer dans le domaine de l'Europe de la défense. Le fonds européen de la défense est une étape vraiment décisive puisqu'il permettra de financer la recherche de défense ainsi que certaines phases de développement de programmes capacitaires,

Le financement partiel du développement de programmes capacitaires est une proposition phare de la Commission qui, au-delà, souhaite pouvoir créer un programme européen de développement industriel de défense. Vous m'avez interrogée sur le calendrier de mise en oeuvre L'objectif est d'adopter le règlement permettant d'engager ces dépenses dans les prochaines semaines ; une réunion aura lieu au mois de novembre à Bruxelles sur cette question. il est envisagé d'affecter 500 millions d'euros en 2019, 500 millions d'euros en 2020, puis, pour les années suivantes, de passer à 1 milliard d'euros par an. évidemment d'être très attentif aux modalités de mise en oeuvre, en vue de nous assurer que les projets financés soient bien définis par les États eux-mêmes. Il faut conclure ! Naturellement- mais il vaut mieux le dire -, ces fonds bénéficient à la base industrielle et technologique de défense européenne.

On y insiste sur la remise en cause des certitudes et le brouillage des lignes, comme le monde en connaît depuis la chute du mur de Berlin. Face à un monde de plus en plus chaotique, complexe et souvent incertain, notre diplomatie a besoin d'un cadre d'action fort, cohérent et ambitieux. Nous avons aujourd'hui le devoir d'oeuvrer en faveur d'un ordre collectif, avec nos alliés et tous nos partenaires. Pour ce faire, la revue préconise plusieurs axes forts pour renouveler la diplomatie de la France une sécurité qui prenne en compte l'émergence de nouveaux acteurs ; une indépendance qui impose de revisiter les termes de la souveraineté, y compris européenne ; enfin, une influence qui va de pair avec la défense des biens communs universels. À cet égard, mon interrogation porte sur l'enjeu que constitue le renseignement économique et financier, sujet actuellement à la croisée de diverses sphères et de plusieurs administrations. En effet, nos impératifs de sécurité nationale s'étendent non seulement à la défense du territoire, mais aussi à la préservation des capacités économiques de la Nation. L'interdépendance et la concurrence économiques à l'échelle mondiale se sont accrues et se révèlent des sources importantes de tensions et de conflits possibles entre les États. L'information s'avère désormais une condition essentielle de la compétitivité. Dans le cadre de la nouvelle loi de programmation militaire, je souhaite connaître les intentions de Mme la ministre des armées concernant le développement de l'intelligence économique, sachant que son importance reste sous-évaluée en France, contrairement à nos partenaires anglo-saxons qui en ont fait une de leurs priorités en matière de renseignement. La parole est

il y va des intérêts du pays. Cette question est à l'intersection de l'action de plusieurs ministères, et le ministère des armées y contribue naturellement. effet, il participe à l'accompagnement des capacités économiques de la Nation. Ce renseignement recouvre différentes thématiques : une thématique politico-économique, une thématique concurrentielle, technologique ou bien financière. Pour ce qui nous concerne, nous nous intéressons à la lutte contre l'ingérence économique extérieure. De ce point de vue, je veux souligner le travail réalisé par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, qui contribue à déceler et neutraliser les menaces affectant le potentiel scientifique et technique de la Nation. Ce combat a enfin une dimension cybernétique, un domaine dans lequel les services de renseignement et l'état-major des armées jouent là encore, aux côtés de l'ANSSI, un rôle central. Vous m'interrogez sur les moyens. Ceux-ci sont en constante augmentation : de 2014 à 2017, les fonctions globalement entendues de cyberdéfense et de renseignement auront vu leurs effectifs augmenter de près de 1 800 emplois. Pour ce qui concerne la seule année 2018, dans le cadre du prochain budget qui sera soumis à votre approbation, ces effectifs augmenteront encore de 848 emplois.

me laisse perplexe sur bien des points, notamment pour ce qui concerne le développement de programmes nucléaires en France. Au-delà du traité de non-prolifération des armes nucléaires, auquel notre pays n'a adhéré qu'en 1992, 122 pays ont adopté en juillet dernier à l'ONU un traité d'interdiction des armes nucléaires. Dans ce contexte, comment expliquer le refus de notre diplomatie de participer aux

Mme la ministre. Madame la sénatrice, le désarmement nucléaire reste un sujet de préoccupation majeur pour notre pays. Il est nécessaire si l'on veut aboutir un jour à un monde sans armes. Ce principe de désarmement est actuellement encadré par un traité de non-prolifération, qui reste aujourd'hui la norme fondamentale en matière de désarmement nucléaire.

qui cherchent à adopter l'arme nucléaire. Il nous semble donc tout à fait prioritaire, essentiel

Au-delà de la menace terroriste, il y a les enjeux migratoires, le contrôle des frontières, la protection des événements sportifs et culturels notamment. L'évolution récente de l'opération Sentinelle semble au final assez homéopathique elle permettra sans doute à l'armée de terre de sortir du sur-régime, mais le totem des 10 000 soldats est toujours là, et l'articulation avec les forces de sécurité intérieure n'est pas repensée en profondeur. La vraie question me semble aller au-delà des effectifs et de l'articulation des différentes forces. Il faut s'interroger sur le rôle même de l'armée en matière de sécurité intérieure. Est-ce, par exemple, à l'armée d'assurer des missions de police aux frontières ? Alors que les forces de police et de gendarmerie sont à bout de souffle après des mois de lutte contre le terrorisme et de maintien de l'ordre, l'armée elle-même extrêmement sollicitée sur les théâtres extérieurs fait office de palliatif. L'opération Sentinelle devait être provisoire, comme, d'ailleurs, l'état d'urgence. On sait aujourd'hui que la menace terroriste ne cesse de se renforcer. Les revers de l'État islamique en Irak et en Syrie font craindre le retour rapide des djihadistes français et de leurs familles, qui cultivent la haine des juifs, des mécréants et de toutes nos valeurs humanistes et républicaines. Ne faut-il pas alors, madame la ministre, repenser complètement le système et clarifier la situation afin de savoir si nos armées doivent se concentrer sur les opérations extérieures ou assurer la sécurité intérieure, à moins que vous ne souhaitiez renforcer considérablement leurs effectifs ? Très bien

Des savoir-faire et des matériels particuliers viennent donc en appui de tous les secouristes, civils ou autres, qui se sont engagés sur ces terrains. De ce point de vue, la présence du bâtiment de projection et de commandement a été un

conférés à l'armée de terre, qui a vu le nombre de ses effectifs progresser de manière importante pour pouvoir répondre à ses besoins.

professionnalisme et protègent la sécurité des Français. Il ne s'agit pas du tout de mélanger les genres. Il faut continuer à entraîner et à maintenir nos soldats

Perrin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la revue stratégique présentée la semaine dernière devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées par Arnaud Danjean est un document « solide », pour paraphraser le président Cambon. Je souhaite Je souhaite remercier et féliciter son auteur, ainsi que le comité de rédaction, de ce travail remarquable : ils ont travaillé vite et bien, ce qui nous permet de nous concentrer sur la loi de programmation militaire sans perdre de temps. Madame la ministre, la revue prône le maintien d'un modèle d'armée complet et équilibré. Entre les menaces diffuses de basse intensité et le retour des États-puissance, il va falloir dessiner des priorités pour nos armées. Dans ce contexte, il s'agit de définir les pays européens volontaires politiquement et, surtout, capables militairement de participer à une coopération. Des choix stratégiques majeurs vont devoir être faits

Se pose aussi la question de la surveillance aérienne du territoire national, qui doit être repensée. La surveillance des frontières ou des grands événements comme les Jeux olympiques de 2024 est à préparer dès maintenant. Les drones sont un nouvel outil à exploiter. Les besoins et les demandes en la matière vont exploser et, tout comme nous ne faisons plus aujourd'hui d'opération militaire sans un drone, sans doute demain n'organiserons-nous plus aucune manifestation ni aucun grand événement sans un drone. Les Harfang seront prochainement retirés du service, les Reaper et les Patroller seront largement, voire exclusivement mobilisés pour les opérations extérieures. La prochaine loi de programmation militaire permettra peut-être- vous nous le direz -de mobiliser de nouveaux moyens de nature à aller dans le sens que je viens d'évoquer. Enfin, quelle étape supplémentaire faut-il franchir pour préparer l'avenir ? Envisagez-vous de passer du drone armé au drone de combat ? Quel sera le système de combat du futur ? La parole est à Mme la ministre.

de réduire les risques encourus par les équipages. J'ai donc fixé trois priorités au ministère des armées. La première consiste à conforter notre capacité d'acquérir du renseignement au moyen de drones aériens. Pour cela, nous allons poursuivre la livraison des systèmes de drones Reaper, mettre en service le système de drones tactiques Patroller et préparer le futur drone MALE européen.

la revue stratégique dresse un tableau global de l'environnement dans lequel notre pays et l'Europe évoluent. Sur ce point, la partie touchant à la sécurité continentale mérite, me semble-t-il, une attention particulière. L'analyse de la « déconstruction de l'architecture de sécurité en Europe » paraît singulièrement juste, au regard notamment des entreprises de déstabilisation engagées par Moscou à l'endroit de l'Ukraine, qui font fi de tous les traités et des fondements les plus élémentaires du droit international. Dans le même temps, force est de constater que l'unilatéralisme dont l'administration Trump se prévaut participe de ce registre et nous touche collectivement en tant qu'Européens. En témoignent ainsi non seulement sa volonté de désengager les États-Unis de la COP 21, qui met en péril l'ambition de réguler le changement climatique, mais également celle de remettre en cause l'accord historique de Vienne sur le nucléaire iranien, alors même que celui-ci a vocation à être un important outil de stabilisation d'une partie du monde pour le moins tourmentée. Cette posture, qui devient une constante de la politique extérieure américaine et qui va à l'encontre des intérêts européens, sur le lien transatlantique, pourtant valorisé par la revue stratégique comme un « élément clé de la sécurité européenne », l'OTAN restant « pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre N'y a-t-il pas, madame la ministre, une contradiction entre, d'une part, la telle valorisation d'une alliance, certes importante au regard de l'histoire et du rôle qu'elle joue mais qui semble tout de même peu ou prou en voie de délitement, et, d'autre part, la volonté de tendre vers « une autonomie stratégique européenne », actée par la revue ? Comment envisagez-vous de concilier le nécessaire développement d'une Europe de la défense avec le maintien de ce lien transatlantique aujourd'hui fortement fragilisé et pour le moins imprévisible ? La parole est à Mme la ministre.

de ce fait, me semble-t-il, une parfaite cohérence entre la démarche que les Européens adoptent dans le cadre de l'Union européenne et ce que l'OTAN

Je ne vois pas de contradiction entre l'un et l'autre ; je vois au contraire un renforcement et des synergies qui vont s'exercer de l'un vers l'autre. En outre, le fait que nous soyons aux avant-postes de la construction de l'Europe de la défense ne signifie nullement que nous nous désengagions en quoi que ce soit de l'alliance sur la frontière estonienne, où nous avons des bataillons engagés aux côtés de bataillons britanniques dans le cadre d'une force de l'OTAN

D'abord, les menaces persistent, voire s'accroissent. Il y a certes des victoires au Levant- saluons le symbole de Raqqa -, mais le Sahel n'est pas stabilisé et Boko Haram reste actif. Qu'adviendra-t-il si les djihadistes chassés du Levant se replient dans cette zone ? La République centrafricaine mais aussi la République démocratique du Congo ne peuvent qu'inspirer de vives inquiétudes ... Ensuite, deuxième impératif, il faut ménager l'outil pour durer, car notre niveau d'engagement est éprouvant pour les hommes et pour le matériel. Cet aspect a été maintes fois souligné. troisième point, il faut chercher des soutiens, en Europe, d'abord, quand nos partenaires ne partagent pas notre priorité sahélienne, aux Nations unies, ensuite, alors que l'attitude des États-Unis a compliqué l'adoption de la résolution 2359 sur la force du G5 au Sahel,

l'autonomie stratégique ne saurait se penser en termes exclusivement militaires et suppose une articulation étroite avec [ ...] [la] diplomatie [ ...] [et le] développement. » Madame la ministre des armées, comment contribuerez-vous à créer, avec M. le ministre des affaires étrangères, une véritable dynamique défense-diplomatie-développement, dans une optique de sortie de crise au Levant et au Sahel, mais aussi dans une perspective préventive dans un Maghreb fragile ?

Nous voyons bien que nos adversaires sont des groupes armés terroristes et que l'action contre de tels groupes ne peut être uniquement militaire ; cela ne serait pas suffisant. Il faut, vous l'avez rappelé, lier de façon cohérente une approche diplomatique et politique- l'engagement opérationnel de nos forces armées -avec une aide au développement qui permet, au fond, de répondre

cette approche globale, qui n'est pas nouvelle. Au sein du ministère des armées, le Centre interarmées des actions sur l'environnement est spécifiquement chargé de contribuer à sa mise en oeuvre, en

Sur le terrain et à l'échelon local, nous mettons également quotidiennement en oeuvre cette approche au travers d'actions civilo-militaires ou de l'aide médicale déployée en faveur des populations partout où nos troupes sont présentes. D'une façon plus ambitieuse, à l'échelon de la région sahélienne, la création de l'alliance pour le Sahel répond également à cette logique.

chers collègues, j'ai le grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation du Sénat du Cambodge, conduite par Mme la présidente de la commission des affaires étrangères et de la coopération internationale du Sénat cambodgien. Cette délégation effectue actuellement un séjour d'étude dans notre pays, notamment sur le thème de la diplomatie parlementaire. Après une journée d'entretiens au Sénat hier, au cours de laquelle elle a été reçue par notre collègue Vincent Éblé, qui préside notre groupe d'amitié la délégation s'est entretenue tout à l'heure avec notre collègue Jérôme Bignon, membre de la délégation du groupe français auprès de l'Union interparlementaire. Elle rencontrera tout à l'heure M. Philippe Mouiller, membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous sommes sensibles à l'intérêt que la délégation porte à notre institution, dans le cadre des relations inscrites dans l'histoire et fructueuses qui existent entre nos deux assemblées. Au nom du Sénat de la République française, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue et je forme des voeux pour que son séjour en France lui soit profitable et contribue à renforcer encore les liens qui unissent nos deux pays. Dans la suite du débat interactif, la parole est

comme nous tous ici, j'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Je veux saluer la qualité du travail réalisé par son comité de rédaction, présidé par notre collègue député européen, Nous ne pouvons que partager le constat d'une France exposée et engagée dans un environnement de plus en plus instable et en proie à des menaces de plus en plus diffuses. Ce contexte périlleux nous oblige plus que jamais à être en capacité d'action et de réaction sur notre territoire national, bien sûr, mais aussi en de nombreux points du globe. Madame la ministre, considérant que cette revue stratégique est le préalable à la préparation d'une nouvelle loi de programmation militaire, je souhaite vous sensibiliser à la nécessité d'envisager d'ores et déjà la construction d'un porte-avions nucléaire à même de succéder au. Véritable Véritable fer de lance de notre capacité de projection et d'intervention lors de situations de crise, le porte-avions constitue une composante majeure de cet « outil de défense agile, projetable et résilient » qu'appelle de ses voeux le Président de la République dans la préface de ce « modèle d'armée complet et équilibré [ ...], le seul à [même de] donner à la France les moyens de son autonomie stratégique et de sa liberté d'action » que vous évoquez vous-même, madame la Il ne s'agit pas d'entrer aujourd'hui dans un débat sur le budget futur des armées, mais bien d'anticiper- près de vingt ans ont séparé les premières études pour la construction du et son admission au service actif en 2001 -, avec cette exigence qui doit être la nôtre : leur donner des moyens opérationnels modernes et maintenir ces moyens à un niveau de performance. Il s'agit aussi de ne pas perdre un savoir-faire technologique et industriel qui a fait ses preuves et de conserver une position forte en matière de défense en Europe, plus particulièrement au sein de l'Union européenne post-Brexit. Enfin, envisager la permanence de cette capacité constituerait un signal fort vis-à-vis de nos armées, dont nous ne saluerons jamais assez le sens du devoir, le professionnalisme et la compétence. Mme la ministre. Monsieur le sénateur, ce modèle d'armée complet que la revue stratégique appelle de ses voeux repose notamment sur la capacité de se projeter depuis la mer. Pour cela, nous disposons déjà de trois bâtiments de projection et de commandement, ou BPC, qui permettent de projeter des troupes, de conduire des opérations amphibies et de projeter outre-mer les moyens de l'État, comme cela s'est récemment fait aux Antilles. Au-delà, la capacité de projection depuis la mer passe aussi par les avions, qui doivent pouvoir décoller d'un porte-avions. La résurgence des États-puissance se traduit en ce moment par la construction de nombreux porte-avions dans le monde en Chine, en Inde ou encore au Royaume-Uni. Ce constat nous rappelle que les porte-avions sont des outils militaires exceptionnels, qui fournissent non seulement une capacité de projection vers la terre mais encore une capacité d'acquisition autonome de renseignement et, surtout, de contrôle des espaces aéromaritimes. Bref, c'est un outil majeur du combat naval.

un vecteur de crédibilité vis-à-vis de nos alliés ; les récentes opérations que nous avons menées en Méditerranée, en lien avec nos alliés américains, en attestent. Dès la prochaine loi de programmation militaire, nous devrons lancer des études pour renouveler cette composante des porte-avions.

qui n'est pas souvent abordée. L'industrie spatiale française bénéficie de nombreux atouts. Elle est l'un des au niveau mondial ; il faut désormais tirer avantage de son excellence pour enraciner dans le paysage industriel français des compétences incomparables tournées vers les besoins du futur, facteurs d'indépendance technologique et de rayonnement politique et stratégique. Comme le précise la revue stratégique de défense et de sécurité nationale, l'espace exoatmosphérique est en profonde mutation et en proie à des logiques de compétition tant militaire que stratégique. Des acteurs étatiques et non étatiques disposent aujourd'hui de moyens industriels leur permettant de mettre en place des satellites. Les prouesses technologiques et scientifiques des dernières années ont contribué à l'essor d'une nouvelle manière de concevoir et d'exploiter les systèmes spatiaux, sur fond de compétition accrue entre acteurs étatiques, sur le plan tant politique qu'industriel. Support de services aujourd'hui indispensables de navigation, de communication, de météorologie ou d'imagerie, le domaine spatial est aussi un espace de confrontation des États peuvent aujourd'hui être à l'initiative de la mise en place de technologies potentiellement antisatellites. Les activités liées à ce nouveau schéma posent également des questions d'ordre juridique. Le problème de l'« arsenalisation » de l'espace se pose donc en des termes renouvelés. Face à ces nombreux défis, nous devons nous doter d'une politique spatiale ambitieuse. Pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, quel pourraient en être les contours dans la prochaine loi de programmation militaire ?

que constitue l'espace en tant qu'espace militaire potentiel, même si la politique spatiale n'est évidemment pas nouvelle, et elle met le doigt sur les menaces que tout cela comprend.

quelques très rares grandes puissances devient aujourd'hui possible pour des entités non étatiques, avec, finalement, peu de moyens. Par ailleurs, vous l'avez souligné,

Nous travaillons par ailleurs à l'introduction d'un certain nombre de systèmes spatiaux dans la prochaine loi de programmation militaire. J'ai participé ce matin à une

La revue stratégique de défense et de sécurité nationale fait le constat inquiétant de la multiplication des menaces non étatiques du fait de la dissémination plus importante des armes. Sous le précédent quinquennat, l'industrie de l'armement servait de variable d'ajustement à notre balance commerciale, c'est du moins notre vision. Madame la ministre, le Gouvernement entend-il revoir notre politique d'exportation d'armement ? La parole est à Mme la ministre. Mme la ministre. Madame la sénatrice, le développement de l'exportation en matière d'armement est un prolongement indispensable du développement de ces programmes eux-mêmes. Aujourd'hui, sans l'exportation, un certain nombre de programmes militaires ne pourraient pas être menés à bien. L'exportation fait donc partie intégrante, en quelque sorte, du modèle de développement de ces programmes.

Il existe des règles internationales que nous respectons, sous la surveillance des entités compétentes.

extérieurs. Deux axes contradictoires ressortent avec force de la revue stratégique : d'une part, des enjeux sécuritaires de première importance- en effet, la menace se renforce, se généralise, se durcit, se complexifie, rendant improbable un reflux des interventions extérieures d'autre part, une concomitance d'opérations et de déploiements dans la durée, qui engendre un phénomène d'usure de nos ressources humaines et matérielles. Les armées françaises ont un grand besoin de se régénérer et le maintien de nos capacités est un véritable défi. Des programmes de renouvellement du matériel ont été engagés ; je pense principalement au programme Scorpion, qui devrait offrir un certain renouvellement des capacités de combat et de soutien de l'armée de terre à moyen terme. En attendant, la situation est particulièrement tendue. L'exemple le plus symptomatique, évoqué par notre président, est celui des véhicules de l'avant blindé. Leur taux de disponibilité est d'à peine plus de 42 %, et leur âge moyen de trente Leurs coûts de maintien opérationnels sont extrêmement importants et les mécaniciens ne pourront pas faire éternellement des miracles. Madame la ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait plus efficace de concentrer les crédits sur un renouvellement accéléré de ces engins, permettrait d'offrir un niveau de protection plus important à nos militaires, plutôt que de subir des coûts extrêmement élevés de maintien en condition opérationnelle ? Cette disponibilité des matériels comporte des dimensions plus globales, c'est la seconde partie de ma question : les opérations extérieures françaises vont-elles être réarticulées en fonction des priorités dégagées par la revue stratégique ?

qui sillonnent les pistes du Sahel et qui sont très exposés à la menace d'engins explosifs. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais il s'agit là de l'une des priorités du prochain projet de loi de finances.

nous ne voyons pas à ce stade de réduction possible à très court terme de nos engagements.

M. Rachel Mazuir. Madame la ministre, la principale nouveauté de la revue stratégique par rapport au Livre blanc de 2013 est la reconnaissance- enfin ! », diront certains -du cyberespace comme un lieu important de conflictualité. La prise en compte des menaces a été amorcée par le développement d'une politique de cybersécurité par l'ANSSI. Sans doute faudra-t-il aller plus loin, compte tenu de l'évolution des menaces qui persistent. Nous savons que le Secrétariat national de la défense et de la sécurité nationale prépare une revue stratégique de cyberdéfense. Il est dommage, de notre point de vue, que ce travail n'ait pas été mené en relation plus étroite avec l'élaboration de la revue stratégique de défense, dont le volet « protection » apparaît dès lors moins, voire insuffisamment développé. La revue préconise le renforcement prioritaire des moyens de défense et le développement de capacités offensives, mais aussi défensives. Elle annonce que « la France a décidé de se doter d'une posture permanente de cybersécurité et va jusqu'à poser le postulat d'une invocation de l'article 51 de la charte des Nations unies dans l'hypothèse d'une cyberattaque, ce qui nous permettrait de riposter sans avoir à attendre l'avis de qui que ce soit. Pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, si le Gouvernement entend remettre en cause le modèle original français de séparation des instances qui sont chargées de la protection et de celles qui s'occupent de la lutte informatique offensive ? informatique offensive, la revue stratégique insiste sur les capacités de détection et d'attribution, c'est-à-dire la recherche des coupables- ce n'est pas le plus facile -, ainsi que sur la capacité pour nos armées de planifier et de conduire les opérations dans l'espace numérique jusqu'au niveau tactique de façon intégrée et d'exploiter ainsi la numérisation croissante de nos adversaires. S'agit-il d'une évolution de cette doctrine ? Enfin, quel format pensez-vous donner au commandement cyber dans le cadre de la loi de programmation militaire ? À combien évaluez-vous le montant des crédits nécessaires pour doter nos armées de capacités crédibles en personnels, bien évidemment- il faut les former -, mais aussi en moyens techniques ? La parole est

Dans le domaine cyber, la mission de renseignement et d'investigation revêt une très grande importance. Elle suppose des moyens dédiés, qui ne sont pas tous de nature numérique. Nous avons en effet besoin de mobiliser l'ensemble de la panoplie, laquelle comprend également le renseignement humain. La deuxième mission de la fonction cyberdéfense, c'est la posture de protection et de défense. Elle intègre une défense en profondeur, qu'on appelle la cyberprotection. consiste à bâtir d'épaisses murailles, ainsi qu'à veiller en permanence à leur efficacité, face à une menace toujours évolutive. La fonction cyberdéfense intègre qui est la lutte informatique défensive. Elle consiste à patrouiller, à guetter et à intervenir dans l'espace numérique en cas d'intrusion pour éradiquer la menace et reconstruire la muraille. Enfin, la troisième mission est la lutte informatique offensive, que je caractériserai par deux termes : riposte et neutralisation. Il y a une distinction entre ce que fait l'ANSSI, qui est focalisée sur les aspects de défense, et ce que font les armées, qui sont centrées sur l'offensive. Cette distinction n'a pour l'instant pas lieu d'être remise en question. La revue stratégique de cyberdéfense va très prochainement rendre ses conclusions.

La revue stratégique se fait l'écho de ces préoccupations. Nombre des technologies disruptives d'intérêt militaire dérivent plus que par le passé, et de façon croissante, de technologies civiles. Ces évolutions sont manifestes dans la sphère numérique. L'hyper-connectivité, les technologies du, l'internet des objets, la robotique, l'utilisation de l'intelligence artificielle vont avoir un impact non seulement sur les armements, mais aussi sur la conduite des opérations de renseignement et de combat. La diffusion de ces technologies efface les écarts de puissance entre États et offre également des capacités à des groupes terroristes ou criminels incontrôlés. Il faudra donc également prémunir nos administrations, nos services publics et, bien sûr, nos armées contre les risques de détournement et de pertes de contrôles de leurs propres systèmes. Comment ces évolutions sont-elles intégrées par nos armées dans leur réflexion doctrinale ? Impliquent-elles de nouveaux modes d'organisation dans la conduite des opérations ? Comment le commandement militaire prépare-t-il ces évolutions et y prépare-t-il les personnels ? Quels projets concrets vont, dans un avenir proche, trouver une application opérationnelle jusqu'au niveau du combattant ? La conduite des programmes d'équipement doit-elle être pensée pour être plus agile, intégrer plus rapidement des technologies dérivées d'applications civiles, voire faire travailler ensemble start-up, officiers de programme et chercheurs sur des projets, tout en préservant nos capacités souveraines ? Un projet comme Intelligence Campus, soutenu par la direction du renseignement militaire, vous paraît-il correspondre à ces nouveaux modes d'organisation ? La parole est à Mme la ministre.

des modes d'innovation différents, à savoir les modes d'innovation qui se développent dans le monde civil, sur des cycles très courts, et les modes d'innovation et de développement technologiques sur des temps plus longs, tels que ceux que nous avons l'habitude de mettre en oeuvre au sein du ministère des armées.

ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème favorable à l'innovation afin de permettre des fertilisations croisées entre le monde civil et le monde militaire. Il s'agit également de permettre l'accélération de l'innovation au profit des armées,

visiter Intelligence Campus, mais ce campus fait partie des sujets dont je vais m'entretenir avec la direction du renseignement militaire. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il

assurer le caractère sûr et opérationnel de nos équipements. Nous devons développer nos outils de simulation

la photo est émouvante : un militaire souriant porte dans ses bras une petite fille endormie. Nous sommes dans l'aérogare de Saint-Martin, l'île ravagée par l'ouragan Irma. Cet instantané, publié par l'envoyé spécial de Radio France, a déclenché une étonnante polémique sur les réseaux d'opération de propagande de l'armée française, de néo-colonialisme ! Il y a quelques jours, un faux sondage circulait par e-mail sur le mode : « saviez-vous que ? » Cette manoeuvre visait à lister les prétendus avantages, aussi faux qu'astronomiques, dont bénéficieraient les sénateurs. Je mesure les efforts entrepris pour nous protéger contre les cyberattaques et ceux qui sont annoncés pour doter nos armées de capacités de lutte informatique offensives, mais ces efforts seront incomplets si nous ne nous préoccupons pas des actions d'influence et de déstabilisation. La revue stratégique relève la perméabilité des sociétés européennes à la propagande djihadiste, laquelle « a fragilisé les sentiments d'appartenance, affectant ainsi la cohésion des sociétés ». Nous sommes également l'objet d'actions conduites par des puissances étatiques de premier rang, dotées d'extraordinaires arsenaux d'influence et de déstabilisation, qui vont de la diffusion massive de à la manipulation des processus électoraux, comme on l'a vu lors de la campagne présidentielle américaine. L'instrumentalisation des réseaux sociaux est désormais considérée par le Pentagone comme la plus grande menace militaire des années à venir dans le domaine des guerres hybrides. Je suis inquiet face à l'absence dans la revue stratégique d'exposé de stratégie de contre-influence et de promotion de nos valeurs démocratiques. Pouvez-vous Pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, les dispositifs d'ores et déjà mis en oeuvre par le Gouvernement dans ce domaine. Quel est le service chargé de lutter contre la propagation de fausses nouvelles ? La parole est à Mme la ministre.

Numérique, robotique, miniaturisation, intelligence artificielle sont autant de défis pour l'avenir de notre défense. L'innovation, avec sa part de risques, doit être placée au coeur de la démarche du ministère des armées. En effet, nous devons considérer que les défaillances d'investissement d'aujourd'hui pourraient être les lacunes capacitaires de demain. La remarque vaut tout autant pour les armements que pour notre analyse stratégique. Or les perspectives que vous présentez font état d'un risque de « décrochage technologique dont notre pays pourrait être victime ». Dans un environnement où le secteur civil produit de plus en plus de technologies d'intérêt militaire, le risque de « nivellement opérationnel » décrit dans votre document existe bien. Aujourd'hui, avec peu de moyens, des forces armées régulières ou irrégulières, voire des groupes terroristes, peuvent mettre en échec ou entraver l'action de nos forces conventionnelles. Cette problématique vitale doit être prise en compte pour le renouvellement de nos systèmes d'armes. Dans ce cadre, le recours à une meilleure synergie entre la recherche civile et le monde militaire peut se révéler extrêmement bénéfique. Madame la ministre, en plus des dispositifs existants, quelles nouvelles mesures prendrez-vous afin d'encourager une forme de symbiose dans le domaine de la recherche ? Quelle sera notre capacité d'investissement à cet effet ? Par ailleurs, une base industrielle et technologique forte est indispensable. La revue stratégique met opportunément l'accent sur ce point. Or son renforcement passe aussi par des consolidations industrielles. En particulier, quel résultat donnera l'accord de principe trouvé à l'occasion du déblocage du dossier STX sur un partenariat structurant dans le secteur de la construction navale ? Peut-on croire à un Airbus des mers militaire, associant Naval Group et Fincantieri ? La parole est à Mme la ministre. Mme la ministre. Monsieur le sénateur, le ministère des armées, en particulier la DGA, dispose d'un certain nombre d'outils pour encourager et soutenir l'innovation.

le dispositif ASTRID, en partenariat avec l'ANR ; le soutien des pôles de compétitivité, un dispositif rapide en faveur de l'innovation des PME ; des contrats d'étude pour préparer les équipements futurs pour un montant de 700 millions d'euros par an

Enfin, vous m'interrogez sur le projet de consolidation entre Naval Group et Fincantieri. Ce projet a été lancé sous forme d'études à conduire lors du précédent sommet franco-italien qui s'est déroulé à Lyon. En ce moment même, les équipes de Fincantieri et de Naval Group, accompagnées par le ministère des armées et le ministère de l'économie de chacun de nos deux pays, travaillent

humaine, matérielle et financière du ministère des armées ? Vous avez annoncé tout à l'heure la trajectoire budgétaire,

Mme la ministre. Monsieur le sénateur, j'ai en effet indiqué que, à partir de 2018, les moyens consacrés au ministère des armées remonteraient en puissance. Cette remontée en puissance était indispensable

Nous devons aussi préparer le futur. La prochaine loi de programmation militaire devra trouver un juste équilibre entre ce qui est absolument indispensable, c'est-à-dire la reconstitution de notre

la préparation de l'avenir, c'est-à-dire de prendre des décisions qui n'auront d'effets visibles, dans certains cas, que dans trente ou quarante ans. Oui, monsieur le sénateur, j'ai conscience

d'aborder deux sujets indissociables. J'évoquerai tout d'abord le rôle de la gendarmerie nationale dans la défense de notre pays, de ses intérêts et de nos ressortissants, tant sur le sol national qu'à des milliers de kilomètres, dans nos territoires ultramarins. On ne peut envisager la doctrine de sécurité sans prendre conscience de la spécificité évidente de la gendarmerie : son ancrage territorial, ses capacités judiciaires, militaires, administratives, ses relations privilégiées avec nos concitoyens et les autres armées. Dans le contexte de menace terroriste, nous ne pouvons ignorer l'aggravation de la porosité entre les activités criminelles et le financement d'organisations djihadistes transnationales. en matière de lutte contre le trafic d'armes en provenance des Balkans occidentaux ou de drogues en provenance de la bande sahélo-saharienne, la gendarmerie a une véritable expertise des filières et de leurs interactions. Madame la ministre, alors que le risque d'attentat ne cesse de croître, dans quelle mesure les métiers de la gendarmerie, qui ont une réelle valeur ajoutée dans notre outil de sécurité nationale, peuvent-ils être optimisés et développés ? Enfin, je ne saurais conclure sans évoquer un point capital de notre politique de défense : nos ressources humaines. Vous aurez beau « cybernétiser » ou moderniser, il n'est point de défense sans ressources humaines. Or nous savons tous que celles-ci sont véritablement épuisées. véritablement épuisées. Ne pensez-vous pas que nos militaires, qui ne sont pas des fonctionnaires comme les autres, du fait même de leur condition militaire vingt-quatre heures sur vingt-quatre, mériteraient une réelle amélioration de leurs conditions de travail et de vie, au sens large du terme ?

est une force armée rattachée au ministère de l'intérieur, qui couvre et incarne l'État sur 95 % de son territoire, au profit de la moitié de la population. Elle constitue une force de continuité et de souveraineté, quelle que soit l'intensité des crises. Les gendarmes ont de remarquables capacités remarquables capacités à mener un certain nombre d'opérations en complément de celles des armées elles-mêmes. La gendarmerie apporte en effet des appuis quantitatifs et qualitatifs essentiels, d'abord par l'existence de gendarmeries spécialisées, ensuite grâce à des missions communes réalisées en métropole- c'est le cas dans le cadre de l'opération Sentinelle ou bien outre-mer, par exemple en Guyane, dans le cadre de l'opération Harpie -, enfin

Elle est un acteur clé de l'anticipation dans le cadre de ses activités de renseignement ; elle est un acteur clé de la résilience de la Nation ; elle est enfin également un acteur clé de la dissuasion. dissuasion. L'interopérabilité et la complémentarité entre la gendarmerie et les armées sont des atouts majeurs pour notre pays. pays. Vous rappelez enfin que, sans les femmes et les hommes de la défense, nos armées ne seraient rien. C'est bien pour cette raison, monsieur le sénateur, que j'ai souhaité pouvoir proposer d'ici à quelques jours jours un plan en faveur des militaires et de leurs familles. Je considère que, sans famille heureuse, il n'y a pas de soldat efficace.

Le président Cambon nous a, non sans humour, parfaitement présenté la situation. La politique du toujours plus loin, toujours plus longtemps et avec toujours n'est plus tenable. Il y va de la sécurité même de nos soldats. La multiplication des OPEX sur des théâtres où les conditions sont difficiles, combinée aux besoins de nos forces de souveraineté, pèse sur l'ensemble de notre appareil de défense. Nos matériels sont plus qu'usés, nos soldats sont fatigués et ont des difficultés à maintenir les niveaux d'entraînement. Certes, des efforts budgétaires ont été engagés pour prendre en compte cette problématique,

Mme la ministre. Monsieur le sénateur, le maintien en condition opérationnelle est une de mes préoccupations majeures- j'avoue, pour être tout à fait franche, qu'elle était aussi celle d'un certain nombre de mes prédécesseurs. Que pouvons-nous faire à très court terme ? Dans la mesure où les matériels sont fortement sollicités, il m'a tout d'abord semblé indispensable, dans le cadre des arbitrages budgétaires qu'il a fallu rendre au sein de l'enveloppe globale

question, comment faire en sorte, au-delà des investissements que je viens de mentionner, que nos matériels soient plus disponibles,

dans de nombreux domaines. Je voudrais saluer ce formidable travail, dont nous sommes nombreux à partager les ambitions, tout en nous interrogeant sur la capacité budgétaire à y répondre, même en tenant compte de la hausse annoncée. Se pose aussi un problème d'articulation de la revue stratégique avec la loi de programmation militaire, articulation qui lui a valu d'être surnommée « la rotule » dans le milieu militaire.

si des pays européens non membres de l'OTAN intègrent l'IEI, l'initiative européenne d'intervention,

Mme la ministre.

L'initiative européenne d'intervention a vocation à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et donc l'ensemble des instruments de politique de sécurité et de défense commune.

la question des cadres institutionnels pour favoriser, et c'est finalement la seule chose qui compte, la construction d'une culture stratégique commune entre Européens.

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. Philippe Bas, auteur de la proposition de loi et de la proposition de loi organique. Madame

Les délais ne cessent de s'allonger. En dix ans, ils sont passés de sept mois et demi à près d'un an pour les tribunaux de grande instance. Dans le même temps, le stock d'affaires en attente a augmenté de plus d'un quart. Or le nombre de magistrats et de greffiers a diminué. Les vacances de postes sont devenues endémiques : actuellement, près de 500 postes de magistrats et 900 postes de greffiers ne sont pas pourvus. Les juridictions sont proches de l'embolie.

à tous les magistrats, aux personnels judiciaires et pénitentiaires, aux avocats et aux auxiliaires de justice dont le dévouement quotidien, dans des conditions difficiles, voire dégradées, fait que la justice est encore rendue dans notre pays. Des millions de Français sont concernés. Pour eux, la justice, ce sont d'abord les litiges relatifs aux loyers, aux crédits à la consommation, aux saisies sur salaire, à la propriété, à l'état civil, au droit du travail, au recouvrement de créances et, bien sûr, aux divorces, à la garde des enfants, aux pensions alimentaires ... À l'égard de tous nos concitoyens en demande de justice, les tribunaux doivent avant tout répondre à des impératifs de service public qualité, facilité d'accès, simplicité de fonctionnement, rapidité et, bien évidemment, effectivité de l'exécution des jugements. Il suffit d'énoncer toutes ces exigences pour mesurer le chemin qui reste à accomplir pour répondre aux attentes des Françaises et des Français. En attestent aussi les lenteurs et les dysfonctionnements de l'aide juridictionnelle, ainsi que l'incroyable complexité du partage des compétences entre tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance. Dans notre pays, le parcours de l'accès au droit demeure trop souvent labyrinthique. Quant à la chaîne pénale, elle se caractérise par un phénomène de saturation qui prend deux formes : 100 000 condamnations à une peine de prison ferme en attente d'exécution ; 70 000 détenus pour 58 000 places en prison- chaque 800 détenus dorment sur un matelas posé à même le sol. C'est dire l'ampleur des défis que doit relever la justice de notre pays pour sortir de la crise dans laquelle un long délaissement l'a plongée. Pendant près d'un an, la mission pluraliste de la commission des lois a entendu au Sénat non loin de 300 personnalités du monde judiciaire et a accompli de nombreux déplacements à travers notre pays pour apprécier concrètement les conditions de fonctionnement de la justice. a rendu son rapport le 4 avril dernier. Nous sommes parvenus à faire émerger ensemble 127 propositions, dont 125 ont fait l'objet d'un accord entre nous. d'un consensus politique, mais aussi d'un large consensus judiciaire. Au cours de notre plongée dans le monde de la justice, jamais ou presque la question du manque d'indépendance n'a spontanément été soulevée, sauf pour la nomination des magistrats du parquet. L'indépendance de la justice est profondément ancrée non seulement dans notre droit, mais aussi dans la culture et les pratiques des magistrats. Elle n'est en rien menacée. C'est pourquoi nous avons concentré nos réflexions et nos propositions sur la question des moyens, de l'organisation et de la gestion des juridictions plutôt que sur la conception de réformes institutionnelles sans portée concrète qui nous auraient enfermés dans des débats idéologiques dépassés ayant trop souvent servi de prétexte à l'inertie. Les propositions de loi qui vous sont présentées sont le fruit de ce travail. Au cours des quinze dernières années, la demande de justice a progressé beaucoup plus vite que les moyens, même si, contrairement aux idées reçues, ceux-ci ont en réalité beaucoup augmenté, passant de 4,5 milliards d'euros en 2002 à 8,5 milliards d'euros en 2017. Mais cet effort s'est révélé très insuffisant compte tenu de l'explosion du nombre des instances. En réalité, la justice a été négligée, sauf, peut-être, durant la période 2002-2007, au cours de laquelle le budget a augmenté de 37 %. Le rythme de la hausse a ensuite été inférieur de moitié. Pourquoi ce ralentissement ? Parce que dès l'été 2002 avait été votée une loi de programmation des moyens de la justice, mise en oeuvre cent jours après l'élection présidentielle. La sincérité de la priorité donnée à la justice avait alors été démontrée avec éclat La véritable épreuve de vérité permettant d'apprécier la volonté politique de redresser la justice est donc bien la capacité à adopter rapidement une loi de programmation liant le Gouvernement et le Parlement dans l'élaboration et l'exécution des lois de finances de tout le quinquennat. La proposition qui vous est présentée vise à augmenter le budget de la justice de 28 % en cinq ans, avec la création de près de 14 000 postes et de 15 000 places de prison, pour atteindre un budget d'environ 11 milliards d'euros en 2022. Cette

Pour atteindre ces objectifs matériels, la croissance du budget de la justice devra s'élever en moyenne à 5 % par an, c'est-à-dire être nettement supérieure à celle du budget 2017 et du projet de budget pour 2018, qui traduisent pourtant une évolution substantielle par rapport aux années précédentes. Il faut, par ailleurs, mettre la justice à l'abri des mesures de mise en réserve et d'annulation de crédits qui provoquent, depuis si longtemps, une gestion erratique des budgets et une exécution chaotique des travaux programmés sans véritablement contribuer à la maîtrise des dépenses publiques. Des dispositions vous sont proposées en ce sens. Madame la garde des sceaux, je suis heureux de voir que le Gouvernement, après tant et tant de rapports, a lancé le mois dernier une réflexion multiforme sur la réforme de la justice. Les cinq groupes de travail devront vous remettre leurs conclusions en janvier prochain. Je veux croire que l'inscription de nos deux propositions de loi à l'ordre du jour du Sénat n'est peut-être pas étrangère au lancement de cette nouvelle réflexion. Mais, si le Gouvernement a posé de bonnes questions, nous espérons avoir déjà formulé les bonnes réponses ! Ce serait une perte de chance pour la justice que de ne pouvoir disposer d'une loi de programmation que dans le courant de l'année 2019, deux ans après l'élection présidentielle. Si nous voulons oeuvrer au redressement de la justice dans l'unité nationale nécessaire, il faut aller vite. C'est pourquoi il est essentiel que la réforme de la justice soit adoptée dès maintenant par le Sénat et qu'elle devienne ensuite, si vous le voulez bien, un instrument entre les mains du Gouvernement

manquée. Le montant des crédits de la justice n'est bien sûr pas seul en cause. Il faut également poser la question, soulevée à de nombreuses reprises par la Cour des comptes, de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion des cours et tribunaux, ainsi que des prisons. Il serait vain, en effet, de déployer de nouveaux moyens sans une transformation profonde de la façon d'utiliser les moyens existants. La réforme sera le corollaire de l'engagement financier de l'État et, en quelque sorte, sa contrepartie. C'est pourquoi les textes qui vous sont soumis proposent des changements profonds. La création d'un tribunal de première instance permettra de créer une unité de gestion des juridictions de proximité en maintenant l'intégralité des implantations actuelles. Le développement massif de la conciliation et de la médiation concentrera le juge sur son office et accélérera le traitement des litiges. La réforme de l'aide juridictionnelle écartera du prétoire les recours manifestement irrecevables et financera l'accès au juge par le rétablissement d'un droit de timbre modique. L'amélioration de la gestion des ressources humaines, en magistrats comme en greffiers, mettra fin aux vacances de poste endémiques qui paralysent tant de petites juridictions déshéritées. Le renforcement de l'équipe du juge juge permettra aux magistrats de se consacrer pleinement à leurs tâches. Je cite encore le renforcement des pouvoirs budgétaires des chefs de juridiction, l'accélération des processus de dématérialisation des procédures, l'exigence d'études d'impact dignes de ce nom et, enfin, la clarification du régime de l'aménagement des peines. Cette dernière mesure est une nécessité pour rétablir la confiance dans la justice pénale. Il n'est compréhensible ni pour les victimes ni pour les condamnés eux-mêmes que des peines de prison ferme allant jusqu'à deux ans ne donnent lieu, en pratique, à aucune incarcération. Si les alternatives à l'emprisonnement, dont l'essor stagne depuis cinq ans, doivent être développées, il importe de sortir de l'ambiguïté actuelle : une peine de prison ferme est une peine de prison ferme ; elle doit être exécutée, ou alors il faut prononcer une autre peine Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l'ambition de ces deux propositions de loi montre l'attachement que le Sénat porte à notre état de droit. Elles reflètent les attentes profondes de tous les Français, et pas seulement celles des serviteurs de la justice. Sur un marché du droit en pleine expansion, les tribunaux n'ont plus de monopole : nous assistons à l'essor de sites internet proposant un éventail de plus en plus large de services de règlement des litiges. Si la justice continuait à dépérir, si le sursaut était encore différé, une justice de substitution, qui risquerait d'être aussi une justice au rabais, pourrait prospérer. Voilà pourquoi, mes chers collègues, il y a urgence à agir pour la sauvegarde et le redressement de notre justice.

terrain, à Brest, à Marseille, à Dijon, à Élancourt, à Viroflay, à Nancy, à Metz, à Riom, à Bordeaux, à la direction des services judiciaires, à Bobigny, à Saint-Lô, à Lille, à Marmande et à Agen. Pourquoi cette énumération ? Pour montrer à quel point la commission a été au plus près de

des réformes d'organisation et de structures, ainsi qu'un rapport annexé précisant, sur la même période, l'ensemble des réformes à mener, qu'elles soient législatives ou réglementaires, concernant l'évolution de l'organisation et les pratiques administratives. La proposition

La progression des crédits de la mission « Justice » de 8,7 milliards d'euros en 2018 à 10,9 milliards en 2022 inclut la création de 15 000 places de prison,

Un dispositif plus précis en matière d'judiciaire et d'encadrement des sites internet est proposé. Il s'agit d'une mesure très importante qui constitue un élément substantiel de modernisation de notre justice et de son accès.

à l'aide judiciaire et, en particulier, le rétablissement de la contribution pour l'aide juridique, à un niveau modique et modulable, de 20 à 50 euros,

d'efficacité et de gestion des flux. Disons les choses telles qu'elles sont : il y a de la quantité ; il faut lui adjoindre désormais de la qualité pour avoir de l'efficacité.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, auteur de ces deux propositions de loin, mon cher collègue corapporteur, mes chers collègues,

Que ces textes soient inscrits à l'ordre du jour du Sénat témoigne, s'il en était besoin, de l'intérêt soutenu et constant porté par la Haute Assemblée à

ces textes se veulent la traduction, constitue un socle important. Il montre que l'objectif d'améliorer le fonctionnement de la justice dépasse largement tous les clivages partisans. Le débat d'aujourd'hui donnera l'occasion à chacun des groupes qui constituent le Sénat de démontrer que l'on peut s'accorder sur des propositions consensuelles en la matière. J'y vois la confirmation que la transformation de la justice ne doit pas seulement relever d'un enjeu idéologique. C'est pour moi une conviction profonde. Qu'on ne s'y trompe pas ! Cela ne signifie pas que je ne suis pas attentive aux impératifs de l'État de droit et que je ne mesure pas les exigences constitutionnelles ou conventionnelles de protection des libertés publiques

que nous soyons parlementaires ou membres de l'exécutif, nous devons aussi apporter à la justice des solutions concrètes, opérationnelles, qui améliorent vraiment les choses, et non pas des idées préconçues

de « moderniser le service public de la justice en innovant et en maîtrisant la révolution numérique », de « rendre l'institution judiciaire plus proche des citoyens », d'« améliorer l'organisation et le fonctionnement des juridictions en première instance et en appel », d'« accroître la maîtrise des dépenses ou, enfin, de « redonner un sens à la peine d'emprisonnement ». Je partage bien entendu toutes ces ambitions et je tiens d'ailleurs à remercier M. le président de la commission des lois d'être venu m'en présenter l'économie et la portée. le rapport de la mission comme dans les deux propositions de loi, l'accent est tout d'abord mis sur les questions budgétaires. Vous avez raison sur ce point, et le Gouvernement sait qu'il est nécessaire de donner, sur la durée, des moyens supplémentaires à la justice. C'est une volonté forte qui a été exprimée par le Président de la République et par le Premier ministre, qui en a fait l'un des points essentiels de son discours de politique générale en juillet dernier. Les paroles se sont traduites en actes actes : le budget du ministère augmentera de près de 4 % en 2018 à périmètre constant. Dans le contexte contraint de nos finances publiques, une telle augmentation est assez significative. La progression sera encore plus rapide dans les années à venir, puisqu'elle devrait s'élever à 4,3 % en 2019 et à 5,1 % en 2020. En trois ans, le budget de la justice augmentera ainsi de près de 900 millions d'euros. L'un de mes prédécesseurs avait fixé l'objectif d'un accroissement d'un milliard d'euros sur l'ensemble du quinquennat. Cet objectif sera donc quasiment sera donc quasiment atteint sur les trois premières années. Sans en tirer gloire, c'est évidemment un motif de satisfaction, car c'est l'assurance que nous pourrons avoir les moyens indispensables pour soutenir les évolutions profondes que nous souhaitons mettre en oeuvre en faveur de la justice.

Depuis plusieurs années, les discours sur la justice portent essentiellement sur des questions de principe et sur des questions budgétaires. Évidemment, ces enjeux sont légitimes et importants. Mais il faut aussi s'interroger sur l'adéquation de de l'organisation de la justice et de ses procédures avec les missions qui nous sont assignées. Je veux traiter ces questions, car les augmentations budgétaires ne seront efficaces que si nous nous lançons dans une transformation en profondeur de notre système.

d'avoir sur ce point une divergence de nature plus méthodologique que principielle. L'article 34 de notre Constitution prévoit que les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Même si rien ne fait naturellement obstacle à ce que le Parlement prenne des initiatives en ce domaine, il me semble logique, sur le plan institutionnel, que que le Gouvernement, qui détermine et conduit la politique de la Nation en application de l'article 20 de la Constitution, soit à l'initiative d'une loi de programmation pour la justice, laquelle traduit une volonté politique et une action dans la continuité.

Plus fondamentalement sans doute, je pense que l'excellente base de travail que constituent les travaux de la commission des lois doit être encore enrichie par les propositions venues des acteurs mêmes de notre justice.

Cependant, j'ai souhaité aller plus loin dans la consultation de celles et ceux qui peuvent être porteurs d'idées nouvelles, efficaces et réalistes, car j'ai la conviction, après quelques mois passés place Vendôme, que ce sont les acteurs au quotidien de la justice qui détiennent les clés de sa transformation. Sans eux, rien n'est possible. Ce sont eux qui peuvent nous apporter les solutions concrètes dont nous avons besoin pour engager les indispensables évolutions. Leur expérience, leur engagement, leur imagination doivent nous être utiles. J'ai rencontré des magistrats et des personnels qui prennent des initiatives, fourmillant d'idées pour améliorer le traitement des dossiers, aller plus vite, mieux accueillir les justiciables

la transformation numérique, la simplification de la procédure pénale, la simplification de la procédure civile, l'adaptation de l'organisation territoriale, le sens et l'efficacité des peines. Chaque chantier est coordonné par deux chefs de file choisis pour leur expérience sur chacun des sujets. Chaque chantier sera mené selon une méthode spécifique, ajustée au mieux aux besoins de l'exercice. Je suis persuadée que la transformation numérique est la première priorité. Le justiciable ne peut plus comprendre que la justice reste à l'écart de l'évolution numérique, qui facilite l'accessibilité et l'efficacité des services publics. Le numérique offre l'opportunité unique de rendre notre justice accessible à chacun très simplement, de rendre des décisions plus plus rapidement, de réduire les distances géographiques, d'introduire de la transparence sur l'avancée des procédures. Vous l'avez, cher Philippe Bas, très bien écrit. Ce sujet irrigue en réalité tout le fonctionnement de la justice. Ainsi, il n'est pas normal que les justiciables ne puissent suivre l'état de leur procédure en ligne, comme cela se fait, toute toute comparaison gardée, devant la juridiction administrative depuis plusieurs années. Il n'est pas normal non plus que l'on ne puisse pas saisir les juridictions en ligne, notamment pour les petits litiges. Enfin, on ne peut accepter que les procédures pénales ne soient pas dématérialisées, de l'enquête jusqu'à l'audience, et que les magistrats et les greffes se trouvent noyés sous le papier. Le plan de transformation numérique doit être ambitieux. Les acteurs de terrain, par leurs exigences, nous aideront à fixer les bonnes priorités. Cette réflexion autour de la numérisation doit aller de pair avec la réforme des procédures civile et pénale. C'est une question de cohérence, puisque le coeur du procès sera, dans un futur proche, je l'espère, constitué d'un dossier numérique. C'est pourquoi nous avons lancé, avec le ministre de l'intérieur, mon collègue Gérard Collomb, un ambitieux chantier d'amélioration et de simplification de la procédure pénale. Nous souhaitons ensemble - j'insiste sur cette volonté commune, concernant notamment la phase de l'enquête - que l'on puisse alléger et rendre plus efficace et plus fluide le travail des enquêteurs, dans le respect des libertés individuelles.

Je souhaite donc que le débat s'engage, pour évaluer l'ensemble des propositions et, surtout, celles qui sont issues des consultations effectuées auprès des professionnels de la justice, mais aussi, pour la partie qui les concerne, auprès des enquêteurs, qu'ils soient policiers ou gendarmes. Il va de soi que ce chantier trouvera sa concrétisation et ses prolongements dans les textes que nous présenterons au printemps. Il en ira de même pour le chantier sur le sens et l'efficacité de la peine. Notre ordre pénal républicain est fondé sur le principe de l'individualisation des peines. Cela doit demeurer ainsi. Mais la réflexion n'a pas encore suffisamment investi le champ de l'exécution des peines. Je suis pourtant convaincue que, ce qui garantit l'efficacité de la répression, c'est le caractère adapté de la peine, mais aussi sa certitude et sa promptitude. Outre un plan de construction de 15 000 nouvelles places de prison, qui traduit un engagement présidentiel et permettra d'assurer la prise en charge des détenus dans des conditions tout à la fois de plus grande sécurité pour la société et de plus grande dignité pour eux, pour eux, une réflexion doit être conduite sur le sens de la peine. Elle devra prendre en compte ses trois dimensions : sécuriser la société, punir le condamné et assurer la réinsertion sociale de ceux qui ont purgé leurs peines. Nous travaillons sur la manière de donner aux magistrats les moyens de prononcer des peines réellement diversifiées, en ne faisant plus de la peine d'emprisonnement la seule peine de référence et en réinscrivant à son côté des peines autonomes, notamment les peines de travaux d'intérêt général et le bracelet électronique pour les courtes peines. Dans le cadre de ce chantier sera évalué notre système d'aménagement et d'exécution des peines, devenu, vous l'avez rappelé, messieurs les rapporteurs, trop complexe. Il faut aussi nous pencher sur le parcours des détenus en détention et l'aménagement des fins de peine. de peine. C'est essentiel pour la prévention de la récidive et la réinsertion des condamnés. Tous ces points se traduiront par des modifications de notre législation. La simplification que j'appelle de mes voeux portera aussi sur la procédure civile. La réforme de la procédure en appel, qui vient d'entrer en vigueur, doit être pleinement assimilée par les acteurs, et il faut se donner le temps d'une première évaluation avant de la retoucher profondément. En revanche, nous pouvons aller plus loin, me semble-t-il, s'agissant de la procédure civile de première instance. Dans le cadre de la dématérialisation, il faut simplifier les règles de saisine du juge et développer puissamment la conciliation et la médiation. Il nous faudra travailler sur la déjudiciarisation d'un certain nombre de procédures, dans le cadre de ce chantier. Je souhaite, entre autres choses, que l'on puisse expertiser l'idée de deux « procédures cibles » - procédure avec avocat et procédure sans avocat -, au sein desquelles viendraient se fondre les particularismes qui distinguent aujourd'hui les contentieux. Il faut aussi que l'on puisse s'interroger sur l'office du juge et le rôle des parties quant à l'objet du litige : faut-il davantage responsabiliser les parties sur la mise en état du dossier ? Faut-il instaurer une obligation pour le juge de soulever d'office un moyen de pur droit ? de pur droit ? Un juge compétent pour soulever d'office les moyens de droit, c'est en effet une piste pour rétablir l'égalité des armes au profit du justiciable qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'assurer une défense de qualité. Je souhaiterais enfin que l'on puisse réfléchir à la revalorisation du rôle du juge de première instance : pour ce faire, faut-il revoir les cas d'ouverture de l'appel ou encore généraliser l'exécution provisoire ? ? Toutes ces questions seront soumises à la réflexion ; nous ne devons omettre aucune piste et n'éluder aucune question pour apporter les bonnes réponses. il reste un dernier chantier, qui n'est pas le moindre, celui de l'adaptation de l'organisation judiciaire. La proposition de loi en discussion un certain nombre de propositions très précises à cet égard. Cette adaptation est une conséquence inéluctable des réformes profondes que je souhaite mener. La simplification et la numérisation des procédures ne peuvent rester sans incidence sur nos modes de fonctionnement et sur notre organisation. Les nouvelles perspectives numériques, notamment, changeront le rapport des justiciables à la justice, mais modifieront aussi profondément le travail de l'ensemble des professions du droit. À mon sens, le n'est pas possible. On ne peut imaginer une transformation de nos procédures et de nos modes de fonctionnement sans une adaptation de notre organisation, avec une seule idée-force : rendre le meilleur service possible au justiciable, car c'est bien lui qui doit être notre préoccupation centrale. Cela signifie en particulier que les exigences qui s'imposent à notre organisation doivent être fondées sur le respect des principes de proximité et d'efficacité.

où les intérêts des uns et des autres se chevauchent, se confrontent, se retrouvent ou divergent parfois profondément. Le point de vue du Sénat, assemblée de la proximité et des territoires, est en la matière tout à fait essentiel, et j'y serai très attentive.

C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que soit menée une mission de concertation avec l'ensemble des parties prenantes - professionnels du droit, magistrats, fonctionnaires, parlementaires et élus locaux - sur les principes qui doivent sous-tendre notre organisation judiciaire, tels que les principes de proximité, de collégialité, de spécialisation et de mise en cohérence avec l'action de l'État. Des Des propositions me seront faites par les chefs de file de ces chantiers au tout début de l'année prochaine. Je veux cependant d'ores et déjà l'indiquer, cette réforme doit se faire en conservant le maillage actuel de nos juridictions, en maintenant les implantations judiciaires existantes. Les adaptations ne se traduiront par la fermeture d'aucun lieu de justice. Très bien et ne m'appuierai sur aucune carte préétablie. Mon projet ne sera pas fondé sur un quelconque schéma arrêté de manière autoritaire et technocratique. L'adaptation de notre réseau ne résultera que de la réflexion qui a déjà été conduite et de la concertation aujourd'hui engagée.

opérationnelles et déclinées selon un calendrier précis, de manière à ce que nous puissions être prêts à présenter au Parlement un projet de loi de programmation pour la justice, qui comprendra des dispositions pénales, dès le printemps prochain. Je souhaite que les résultats de ces chantiers puissent être restitués dans un cadre législatif avec la plus grande cohérence, car, si j'ai fait le choix de lancer simultanément ces cinq chantiers, c'est parce que j'ai la conviction que la transformation de la justice ne ne pourra résulter que d'une action globale. C'est finalement à cette conclusion que votre commission des lois a également abouti. Sur le fond, des points de convergence existent entre nous, et c'est heureux, que ce soit sur des objectifs généraux ou sur des mesures concrètes. Je pense notamment aux services de communication en ligne fournissant des prestations juridiques ou aux amendes civiles pour les appels abusifs. Sur d'autres points, nous avons des divergences. Je pense au rétablissement en l'état de la contribution pour l'aide juridique ou aux dispositifs qui pourraient rigidifier excessivement la gestion des ressources humaines. Enfin, nombre des questions que vous avez soulevées sont liées aux conclusions des chantiers de la justice que je viens d'engager. C'est le cas concernant les moyens et les effectifs programmés.

Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement est très ouvert et très attentif aux propositions de votre commission des lois et de votre assemblée. C'est une remarquable base de départ, qui alimentera notre réflexion, parallèlement aux consultations de terrain lancées dans le cadre des chantiers de la justice. Si vous le souhaitez, je tiens à votre disposition les questionnaires qui ont été adressés aux acteurs de terrain dans ce cadre. Les contributions de chacun

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la ministre, mes chers collègues, ces deux propositions de loi font suite aux travaux de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice que présidait Philippe Bas. Les travaux de cette mission, qui comportait un représentant de chaque groupe parlementaire, ont donné lieu à un rapport présenté le 4 avril dernier. Ces deux textes partent du constat que la hausse des moyens dévolus à la justice, milliards à 8,5 milliards d'euros entre 2002 et 2017, n'a pas apporté d'améliorations significatives. Trop de réformes sont venues rendre toujours plus complexe le fonctionnement de la justice, tandis que, dans le même temps, l'activité juridictionnelle n'a cessé de croître. Par ailleurs, notre système judiciaire apparaît bien moins classé que d'autres systèmes judiciaires européens. En effet, depuis plusieurs années, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, instance du Conseil de l'Europe créée pour évaluer l'efficacité des systèmes judiciaires, fait le constat d'une relative modestie du budget de la justice française. Selon son rapport, le montant annuel du budget par habitant affecté au système judiciaire est assez faible puisque la France n'y consacre que 64 euros en moyenne, ce qui la place assez loin du niveau de dépenses consenti par des pays dont les structures sont comparables, comme l'Autriche- 96 euros par habitant -, la Belgique- 85 euros -ou l'Italie- 73 euros. Si l'on rapproche le niveau de dépenses pour la justice du produit intérieur brut par habitant, qui est un bon indicateur de comparaison en zone euro, à niveau de richesse comparable, les Pays-Bas réalisent un effort budgétaire presque deux fois plus important que la France en faveur de leur système judiciaire. Outre le fait que le système judiciaire français est moins bien classé que ses homologues européens, les prisons françaises souffrent depuis de nombreuses années d'une situation chronique de surpopulation carcérale. En tant que rapporteur pour avis sur les crédits du programme « Administration pénitentiaire », je souhaite aborder ce problème. Au 1 mars 2017, le nombre de personnes écrouées détenues s'élevait à 69 430 contre 67 580 au 1 mars 2016, soit une augmentation de 2,7 % en un an. Cette augmentation de la population carcérale s'inscrit dans une tendance constante d'accroissement depuis 2000, qui peut s'expliquer par trois facteurs : la suppression des grâces présidentielles collectives, l'augmentation du nombre de condamnations à des peines de prison ferme et l'allongement de la durée des peines prononcées. La surpopulation carcérale est un facteur aggravant des conditions de travail de l'administration pénitentiaire. Exacerbant les tensions, elle peut nourrir des actes de violence à l'encontre du personnel. En 2015, le personnel pénitentiaire a été victime de 4 070 agressions physiques et de 16 040 agressions verbales ; 8 425 agressions physiques entre codétenus et 113 suicides en détention sont également à déplorer la même année. Aussi la situation actuelle de surpopulation dans les prisons françaises nécessite-t-elle une augmentation considérable et une diversification du nombre de places dans les établissements pour assurer aux détenus des conditions d'hébergement dignes et pour améliorer les conditions de travail des agents de l'administration pénitentiaire. En effet, l'augmentation substantielle de la capacité du parc carcéral apparaît nécessaire pour garantir une réponse pénale plus crédible : il est inconcevable que l'exécution des peines soit retardée en raison de la saturation des établissements pour peine. Il est tout aussi contestable que des prévenus, détenus « provisoires » qui bénéficient de la présomption d'innocence, soient incarcérés dans des conditions indignes en maison d'arrêt. La prison doit jouer un double rôle de punition et de réinsertion. Il est donc nécessaire de disposer d'établissements pénitentiaires offrant des conditions matérielles propices à la prévention de la récidive, mais également d'établissements très sécurisés pour les détenus les plus dangereux, notamment ceux Un autre problème auquel il faut remédier sans tarder est l'effectivité de la peine. S'il est certes exagéré d'affirmer que les condamnations à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à deux ans ne sont pas du tout exécutées, toutefois que si le condamné n'est pas déjà incarcéré aucune condamnation à une peine inférieure à deux ans d'emprisonnement ne sera réellement exécutée en établissement pénitentiaire pour toute la durée prononcée par la juridiction. Le fait qu'une personne condamnée semble ne pas subir de sanction pose problème : cette situation jette un lourd discrédit sur notre justice et suscite l'incompréhension des citoyens. pourquoi il apparaît intéressant que le juge de l'application des peines dispose d'un éventail d'alternatives à l'emprisonnement, comme les travaux d'intérêt général. Pour conclure, madame la ministre, notre institution judiciaire a besoin à la fois de crédits et de réformes, et il y a urgence

Depuis des décennies, une lente dégradation des conditions matérielles de l'exercice de la justice est à l'oeuvre dans notre pays, produisant pourtant de rares élans de manifestation, probablement en raison de la retenue naturelle qui caractérise les hommes de robe. Il serait pourtant naïf de considérer que cette dégradation, au prétexte qu'elle serait tue, ne serait pas perçue par nos concitoyens. Cependant, malgré leur lenteur et leur manque de moyens, nos juridictions bénéficient encore, heureusement, de la confiance des Français. Nos tribunaux exercent toujours cette fascination que décrivait Gide dans ses voilà plus de cent ans. Sans doute, beaucoup de justiciables ont été rassurés d'observer comme lui « la conscience avec laquelle chacun, tant juges qu'avocats et jurés, s'acquittait de ses fonctions ». ». La vigueur du sentiment de justice de nos concitoyens dépend en effet essentiellement du grand professionnalisme et du dévouement de l'ensemble des corps du ministère de la justice, lesquels font fonctionner nos juridictions avec des moyens, il faut l'avouer, bien inférieurs à ceux de nos voisins européens. C'est pourquoi nous souscrivons à la démarche du président Philippe Bas lorsque, au moment de réformer, il choisit de se placer à la hauteur des hommes qui rendent la justice, avec la ferme volonté de résoudre leurs difficultés concrètes. C'est le cas, par exemple, au travers de l'article 25 de la proposition de loi, qui vise à permettre à la cour d'assises, statuant en appel, de ne pas réexaminer l'intégralité de l'affaire à la demande du condamné ou du ministère public. Nous croyons fondamental, comme lui, de stabiliser la nomination des magistrats dans une même juridiction au moins trois ans et, pour la préservation de l'expertise acquise, de maintenir dans une même fonction les juges pour la même durée de trois ans. De la même manière, la réforme de l'aide juridictionnelle associant les avocats en amont de l'attribution de l'aide par le bureau d'aide juridictionnelle nous semble aller dans le bon sens. La maîtrise des frais de justice ne sera efficace que si elle repose sur une démarche inclusive, en associant tous les acteurs en présence. Il est indéniable que la réforme passe également par la résolution des difficultés que rencontrent plusieurs avocats. Dans un climat concurrentiel aiguisé par l'augmentation du nombre de confrères, le risque de la tentation d'alimenter les contentieux n'est pas inexistant. Aussi, en parallèle d'une réflexion sur l'établissement d'un à l'entrée dans la profession, cette dernière doit-elle également être protégée de la concurrence déloyale des sites d'information en ligne, qui sont en plein essor. Certaines dispositions de la proposition de loi nous permettront peut-être d'avancer dans ce sens. Si les nouvelles technologies peuvent faciliter le suivi des dossiers et accélérer les délais d'instruction, nous considérons, en revanche, qu'aucune innovation ne pourra remplacer la vertu cathartique du procès.

N'est-ce pas le sens de l'établissement d'amendes extrêmement dissuasives en cas de requêtes abusives ? Mais nous savons que l'abus est difficile à caractériser à l'aune du droit d'ester en justice, qui est une liberté fondamentale. Il sera donc difficile d'asseoir ce principe. En second lieu, il peut paraître inéquitable d'établir un coût élevé pour le pourvoi en rendant l'assistance par un avocat aux conseils obligatoire ; mais saisir la plus haute juridiction, qui ne statue que sur l'application du droit, nécessite l'assistance d'un juriste confirmé pour éviter les saisines inutiles. Là aussi, nous savons que ce combat de surcoût est vain. En outre, au regard de l'obsolescence des outils bureautiques et des moyens de communication internes aux juridictions, il serait incompréhensible d'accorder de si précieux crédits à la construction d'un nouveau site internet ou au développement d'outils de justice prédictive alors qu'il nous faut nous concentrer d'abord sur la justice effective La Convention européenne des droits de l'homme, dans le premier alinéa de son article 6, fait référence au droit qu'a toute personne « à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». C'est le sens du droit au procès équitable. Sur la conciliation, montrons-nous modernes ! Cela peut être vraiment efficace si nous lui donnons une force exécutoire qui engage les parties. La conciliation peut responsabiliser le citoyen tout en permettant d'instaurer un échange, de retisser du lien social et de promouvoir l'idée d'un « vivre ensemble », tout en garantissant la fin du litige. Il faut cependant assurer et rassurer le citoyen sur l'exécution effective de la solution obtenue par la conciliation. Si nous décidons de la rendre obligatoire, il faut engager une homologation judiciaire. judiciaire. La création d'un tribunal de première instance unique par département est un point qui nous paraît secondaire compte tenu de la nécessaire proximité que les justiciables sont en droit d'attendre. Les tribunaux d'instance remplissent aujourd'hui avec brio leur rôle de juge de proximité et tous les acteurs contestent l'existence de sureffectifs perdus dans les méandres de la carte judiciaire. Alors oui, qui trop embrasse mal étreint ! Selon nous, ces textes de programmation auraient gagné à se concentrer sur quelques objectifs prioritaires : l'exécution des peines, la justice familiale et les nécessaires réformes du conseil de prud'hommes et du tribunal de commerce. Cependant, l'exercice a le mérite d'exister et de faire référence. En conclusion, nous sommes tous d'accord pour affirmer que l'humain demeure la matière première de la justice. Le groupe du RDSE espérait que l'augmentation des effectifs affectés aux juridictions serait plus importante. Comme depuis trop longtemps maintenant, l'administration pénitentiaire absorbe la plus grosse part des crédits la première véritable réforme ambitieuse de la justice serait-elle de désolidariser les budgets de l'autorité judiciaire et de l'institution pénitentiaire, ce qui permettrait de distinguer la crise juridictionnelle de la crise carcérale,

organique, pour le redressement de la justice, toutes deux présentées par le président de la commission des lois, M. Philippe Bas. Ces deux textes sont la traduction législative de 42 des 127 propositions formulées

Pendant neuf mois, la mission que vous avez conduite, monsieur Bas, a abattu un travail considérable en effectuant de nombreux déplacements et en procédant à de multiples auditions. Partant d'un constat alarmant, unanime et sans appel relevant combien la complexité et la lenteur de notre système judiciaire contribuent à rendre la justice illisible, vous soumettez à notre assemblée dans ces deux textes des propositions fort intéressantes. Je pense, notamment, à l'amélioration de l'organisation juridictionnelle en première instance et en appel, ou encore à la révolution numérique. Les objectifs affichés de maîtrise des délais, de qualité des décisions rendues, de proximité ou encore d'effectivité de l'exécution des peines sont éminemment importants. Cependant, je m'interroge sur l'opportunité de voter ces textes à la veille de l'examen du projet de loi de finances et à l'orée de chantiers gouvernementaux sur la justice. En effet, la proposition n° 126 du rapport d'information, qui a inspiré les deux propositions de loi, préconisait la présentation au début de la prochaine législature d'un projet de loi de programmation sur cinq ans pour le redressement des crédits et des effectifs, ainsi que des réformes d'organisation et de fonctionnement de la justice. justice. Le 4 juillet dernier, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, répondait, avant le dépôt deux semaines plus tard de ces deux propositions de loi, à cette demande en annonçant l'examen par le Parlement au au premier trimestre 2018 d'une loi quinquennale de programmation des moyens de la justice, laquelle engagera notamment un vaste mouvement de dématérialisation, de simplification et de réorganisation de notre système judiciaire. Le Gouvernement entendait ainsi démontrer sa volonté de faire de la justice une priorité. C'est également la raison pour laquelle les crédits qui lui seront alloués dans le projet de loi de finances que nous nous apprêtons à discuter augmenteront de 3,9 % en 2018 par rapport à l'année précédente, cela dans un contexte général de redressement des comptes publics. Cette hausse budgétaire doit être considérée comme une première étape, puisque la future loi de programmation quinquennale, qui sera examinée début 2018, prévoira de nouvelles augmentations de 4,3 % en 2019 et de 5,1 % en 2020. Par ailleurs, le 6 octobre dernier, vous engagiez, madame la garde des sceaux, un long et exhaustif travail de concertation avec les professionnels de la justice pour faire remonter les attentes et les initiatives innovantes des différents acteurs du monde de la justice, notamment autour des cinq chantiers que vous avez rappelés, à savoir : une transformation numérique de notre justice, qui permettra notamment de faciliter les procédures en ligne des justiciables ; l'amélioration et la simplification de la procédure pénale l'amélioration et la simplification de la procédure civile ; l'adaptation de l'organisation judiciaire ; enfin, le sens et l'efficacité des peines. Les conclusions de ces travaux seront remises en janvier prochain seront intégrées dans ce projet de loi de programmation pour la justice et au sein des projets de loi de simplification civile et pénale qui nous seront présentés au premier semestre 2018. Aussi me semble-t-il judicieux d'attendre, d'autant que le rétablissement dans la proposition de loi de la contribution pour l'aide juridique ou encore l'extension du suivi socio-judiciaire à tous les délits et les crimes font partie des points de divergence qui, à tout le moins, nécessitent de recueillir au préalable le fruit des consultations lancées début octobre. Il ne fait aucun doute que nous avons tous ici conscience de la situation de quasi-misère dans laquelle se trouve l'institution judiciaire, et nous mesurons l'état d'épuisement des magistrats et des fonctionnaires. Notre volonté est évidemment d'oeuvrer pour l'amélioration du fonctionnement de notre justice. Il y va de l'intérêt de tous, professionnels du droit et justiciables, de pouvoir bénéficier d'une justice de qualité. Cette préoccupation dépasse largement les clivages partisans. Néanmoins, parce que je crois sincèrement que le texte de programmation à venir ira dans le sens d'un redressement de la justice, souhaité par tous, et malgré l'intérêt et la qualité des dispositions qui nous sont présentées, lesquelles, j'en suis certain, viendront nourrir le texte gouvernemental, le groupe La République En Marche s'abstiendra de voter ces propositions de loi.

mes chers collègues, bien évidemment, nous partageons le constat initial à l'origine de ces propositions de loi : il est nécessaire et urgent de redresser notre justice, il va de soi qu'il est primordial de sanctuariser le budget de l'autorité judiciaire, comme le prévoit l'article 1 de la proposition de loi ordinaire. Certes, les moyens de la justice connaissent une hausse régulière depuis 2002. Pour autant, selon nous, mais c'est aussi l'avis de nombre d'acteurs du secteur, le budget de la justice n'échappe pas aux logiques d'austérité. Globalement, les moyens qui sont alloués à cette mission, année après année, ne suffisent pas à permettre aux services de fonctionner convenablement. Cependant une question que mon collègue Pierre-Yves Collombat a soulevée en commission des lois comment lire le débat d'aujourd'hui au regard de la Constitution et de son article 40 ? L'idée que ces textes ne fixent que des cadres et ne sont donc pas contraignants

Qu'en est-il exactement, messieurs les rapporteurs ? Par ailleurs, sur le fond, si nous partageons l'objectif de redressement budgétaire pour la justice, nous sommes au regret de constater que l'augmentation des crédits proposée s'inscrit dans la même orientation que celle de ces dernières années : une progression de 5 % par an bénéficiera

Il n'est pas vrai que le texte a été adopté dans un « esprit consensuel », comme l'avance la commission des lois, tout simplement parce que ce texte est loin d'être consensuel et qu'il porte en lui une vision de la société qui n'est pas la nôtre. Six minutes pour évoquer un sujet si important et des propositions si nombreuses sont bien dérisoires ; je me limiterai donc aux points les plus problématiques à mes yeux et à ceux de mes collègues du groupe CRCE. D'abord, je note une grande contradiction dans les propositions avancées : monsieur Bas, vous invoquez plus de proximité et d'accessibilité pour les justiciables. Cependant, dans le même temps, vous souhaitez fermer des lieux de justice, avec la création des TPI, vous voulez faire contribuer les justiciables aux dépenses de la justice, avec le retour du droit de timbre, et vous désirez ajouter des obstacles à l'obtention de l'aide juridictionnelle pour les plus précaires, avec la consultation obligatoire d'un avocat avant toute demande ! La création des tribunaux uniques de première instance ainsi que des chambres détachées n'est pas une bonne chose.

l'exigence de proximité pour les justiciables. La proximité ne doit pas s'arrêter à la première instance, au juge de proximité ou au conseil de prud'hommes, il faut aussi qu'elle demeure au deuxième degré de juridiction. Trouvez-vous satisfaisant pour notre justice qu'un justiciable puisse se retrouver à quatre heures de sa cour d'appel ? l'aide juridictionnelle, le fait de prévoir que toute demande doit être précédée de la consultation d'un avocat ajoute un obstacle supplémentaire au parcours du justiciable qui souhaite saisir la justice et qui n'en a pas les moyens.

Le rétablissement du droit de timbre va, hélas ! dans le même sens. Instaurée en 2011 et supprimée en 2014, cette taxe présentée comme devant aider au financement de l'aide juridictionnelle aura surtout eu pour conséquence de finir de décourager bien des justiciables aux revenus modestes. Pourquoi alors vouloir la rétablir ? Comme ma collègue Cécile Cukierman l'indiquait dans sa contribution au rapport de la mission qui a précédé ce texte, s'attaquer à l'aide juridictionnelle, c'est s'attaquer à la fonction essentielle de la justice, qui est de rétablir l'égalité des armes entre les parties. L'aide juridictionnelle est le moyen précieux d'accéder à la même justice pour tous. En matière de justice pénale, vos propositions nous inquiètent et témoignent de l'urgence qu'il y a à réfléchir sérieusement sur le sens de la peine. Je vous rappelle, mes chers collègues, que celle-ci a trois vocations : punir, protéger la société et réinsérer. Avec ce texte, la réinsertion n'a aucune place ; au contraire, la peine n'est envisagée que sous l'angle de la punition. En outre, l'unique peine considérée comme possible, voire efficace, est la peine de prison.

C'est aussi ce que relève l'Observatoire international des prisons. C'est pourquoi nous demanderons la suppression de l'article 27, car il est essentiel que le juge de l'application des peines intervienne dans tous les cas, le but étant que la peine soit la plus adaptée possible, et ainsi la plus efficace, avec des « projets de sortie » au cas par cas pour une réinsertion réussie. Nous avancerons nos propositions en ce sens lorsque sera examiné le projet du Gouvernement. À cet égard, nous formons le voeu que les chantiers que vous lancez, madame la garde des sceaux, ou qui sont en cours aboutissent à un texte sous-tendu par une tout autre logique- les premières annonces cependant un peu sceptiques ... -, car il y a urgence à prôner et à ériger une justice plus sociale et humaine. Sans cela, toute tentative de redressement sera vaine. La justice fait l'objet d'une politique publique bien particulière, car elle est essentielle à notre État de droit elle ne fonctionne pas bien, c'est toute la société qui s'effondre ... Pour toutes ces raisons, et également parce que la commission des lois n'a modifié leur texte qu'à la marge, sans rien changer à l'économie générale, nous voterons contre ces deux propositions de loi.